J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la mission d'information sur le développement de l'herboristerie et des plantes médicinales, des filières et métiers d'avenir a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l'examen de l'article 10.

en l'état actuel du texte, pourront associer, si elles le souhaitent, les autres collectivités territoriales lorsqu'elles réaliseront des actions d'information sur les métiers et les formations, c'est-à-dire dans le cadre de leurs compétences. Cette faculté permettra aux régions de choisir les acteurs du territoire utiles et pertinents selon le type d'actions réalisées, qu'elles soient organisées en établissement scolaire ou ailleurs. Inscrire cette obligation d'association des autres collectivités dans la loi pourrait créer des contraintes excessives pour les régions

très intéressés par les métiers du numérique. Pourtant, c'est un secteur d'avenir, désormais incontournable et qui offre d'innombrables débouchés. Je voudrais citer le chiffre suivant : rien qu'en Île-de-France, 50 000 emplois ne seraient pas pourvus dans les

l'avis de la commission ? Les régions pourront sensibiliser les élèves et les étudiants aux métiers du numérique lorsqu'elles réaliseront des actions d'information sur les métiers dans les établissements scolaires. Compte tenu de l'émergence de ces métiers et de la forte création d'emplois dans ce secteur, les actions d'information et d'orientation s'adapteront nécessairement à ces évolutions.

Daniel Chasseing. Cet amendement tend à associer les branches dans la détermination des besoins des entreprises, en lien avec les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation, les OREF. Le projet de loi confie l'orientation aux régions. Or, pour aboutir à une orientation répondant aux besoins des entreprises, les régions doivent détenir l'ensemble des informations relatives aux secteurs économiques. À cette fin, les branches professionnelles établissent des analyses prospectives territoriales sur les métiers et les qualifications, réalisées par les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, les OPMQ. Par ailleurs, les OREF peuvent aussi Par ailleurs, les OREF peuvent aussi apporter une contribution. Aussi, il apparaît nécessaire de préciser que le service public de l'orientation doit disposer des informations dont disposent les OPMQ et les OREF. Quel

des rôles respectifs de l'État et des régions pour la réalisation des actions d'information dans les établissements scolaires et universitaires. L'intervention des entreprises et des observatoires régionaux de l'emploi et de la formation dans l'élaboration de ce cadre n'apparaît pas nécessaire. Toutefois, ces actions régionales pourront associer les entreprises, comme c'est le cas lors des forums des métiers et de toutes les opérations territoriales.

Cet amendement a pour objet de donner aux régions les moyens d'exercer leur nouvelle mission d'organisation d'actions d'information sur les métiers et les formations, prévue par le projet de loi. Il a pour objet de faire explicitement reconnaître ces nouvelles missions comme un transfert de compétences, ce qui reste incertain dans la rédaction actuelle. ? Cet amendement est satisfait. L'alinéa 37 de l'article 10 prévoit en effet que les transferts de compétences à titre définitif prévus par cette loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées

les régions doivent pouvoir s'appuyer sur des données précises et exhaustives quant à la situation de l'emploi sur leur propre territoire. C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit de mettre à disposition des régions les observatoires des branches professionnelles dont la finalité est d'accompagner les entreprises

mais il y a tout de même une réalité dans le texte que nous examinons. Les régions récupèrent les missions et les agents des DRONISEP, afin d'élaborer les publications sur l'orientation à visée régionale et d'identifier les filières et les besoins en compétences sur le territoire. Elles pourront, en outre, solliciter les entreprises et les branches professionnelles pour recueillir leurs besoins en emplois et identifier les filières en émergence, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi.

Si l'article 10 transfère aux régions les missions des délégations régionales de l'ONISEP pour les publications de portée régionale, l'Office restera toutefois un établissement public de l'État, qui éditera notamment les contenus de portée nationale concernant l'orientation. Depuis la loi du 5 mars 2014, l'article L. 313-6 du code de l'éducation prévoit que les régions sont représentées au conseil d'administration de l'ONISEP. Toutefois, le décret d'application

Monsieur le ministre,

bénéficient, eux aussi, de la documentation élaborée par l'ONISEP, qui est nécessaire pour leur orientation scolaire et professionnelle. Jusqu'à présent, les élèves scolarisés dans les lycées français à l'étranger ne sont pas mentionnés dans l'article L. 313-6 du code de l'éducation, qui traite de l'orientation scolaire. Pourtant, pour les élèves de ces établissements situés à l'étranger, il est encore plus nécessaire de bénéficier de la documentation fournie par l'ONISEP, compte tenu de la distance géographique qui les sépare des universités et écoles situées sur le territoire français. Cette documentation est d'autant plus nécessaire que ces élèves, contrairement à leurs camarades basés en France, ne peuvent qu'en de très rares occasions assister aux traditionnelles journées portes ouvertes organisées par les écoles, qui peuvent s'avérer décisives dans le choix d'une orientation.

toute connaissance de cause leur avenir professionnel. L'orientation dispensée durant le second degré, on le sait, est capitale pour la réussite des élèves et permet de réduire le taux d'échec dans l'enseignement supérieur. Alors que la question de l'orientation émerge à partir de la seconde moitié du collège et en fonction des notes générales, plutôt que des aspirations, il convient d'informer les élèves des choix qu'ils devront formuler le plus tôt possible, en expliquant clairement et concrètement les formations. Le bloc de quatre années de collège permet de dégager des moments pour que l'ensemble des formations soit présenté aux élèves dès la rentrée en première année, soit en sixième. La perception de certaines orientations repose aussi sur des, qui se forment,

un sondage de l'Institut Montaigne, 81 % des parents d'élèves interrogés estiment que l'apprentissage est un moyen de trouver rapidement un emploi, mais moins d'un parent sur deux l'envisage pour son enfant

Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs ont tenté d'appuyer l'apprentissage avec des allégements de cotisations, des crédits d'impôt et des primes, mais, en définitive, les effectifs n'ont pas été multipliés. Pensons par exemple à l'échec du précédent gouvernement qui, en 2014, se fixait l'objectif de 500 000 apprentis

l'article L. 331-7 du code de l'éducation prévoit déjà qu'un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève aux différentes étapes de sa scolarité du second degré. L'article 10 prévoit également que les régions disposeront d'au moins vingt heures dans le temps scolaire pour informer les élèves de quatrième et de troisième sur les métiers et les formations. Je le répète, la présentation des caractéristiques de chaque formation dès la classe de sixième risque de constituer une exigence supplémentaire assez lourde à réaliser dans le temps scolaire.

sociales approuve le dispositif visant à préparer les élèves de collège à la voie professionnelle et à l'apprentissage par des enseignements dédiés et des stages. Ce dispositif fonctionne bien dans le cadre des classes de troisième dites « prépa-pro ». Nous avons simplement un doute sur l'articulation de ce dispositif, qui serait étendu à la classe de avec celui des classes « prépa-métiers », dont nous avons parlé tout à l'heure. Il conviendrait de préciser la complémentarité et la portée de ces deux dispositifs, mais sur le fond, la commission approuve le renforcement des mesures visant à sensibiliser les élèves au monde professionnel.

En réalité, dans le cadre du parcours défini à l'article L. 331-7 du code de l'éducation, des actions de découverte du monde économique et professionnel sont déjà proposées à tous les élèves de la classe de sixième à celle de terminale.

rectifié. Depuis 2011, la loi permet aux scolaires de réaliser des périodes d'observation en milieu professionnel d'une semaine durant leurs vacances, afin de les aider dans l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Ces stages, dont l'initiative revient aux familles, sont mis en oeuvre avec l'appui des chambres consulaires et rencontrent un vif succès auprès des jeunes et des entreprises, qui plébiscitent cet outil pour aider les jeunes dans la construction de leur orientation. Toutefois, les étudiants ne peuvent bénéficier de cette possibilité, alors même qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se réorienter en cours d'année universitaire et que leur projet d'orientation professionnelle reste bien souvent à définir ou à confirmer. Cet amendement a donc pour objet d'ouvrir la possibilité de recourir aux stages prévus à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation aux étudiants inscrits dans un cursus d'enseignement supérieur.

aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Rien n'empêche qu'une période de stage se déroule pendant les vacances universitaires. Les étudiants, qui sont majeurs pour la plupart d'entre eux ou ont plus de 16 ans, peuvent aussi être employés en CDD pendant leurs vacances, afin d'acquérir une expérience professionnelle. choses sont différentes pour les mineurs. Il apparaît donc peu opportun d'appliquer un dispositif réservé aux élèves à des étudiants, qui ont d'autres possibilités de découvrir le monde professionnel.

? Le renforcement de la découverte du monde professionnel pourra se faire utilement par les dispositifs des classes « prépa-métiers » ou « prépa-pro outre, cette période d'observation d'une journée, qui plus est sur le temps scolaire, présente un intérêt limité, ainsi que le risque d'être rarement utilisée par les élèves, notamment pour des raisons pratiques.

Morin-Desailly. Lorsqu'elle a examiné l'article 10 du projet de loi, la commission des affaires sociales a adopté un amendement de la commission de la culture, saisie pour avis, visant à renforcer la formation des enseignants aux professions et aux métiers. Je partage bien entendu la volonté exprimée par les rapporteurs de prévoir que les enseignants, les personnels d'inspection et les chefs d'établissement de l'éducation nationale puissent bénéficier, dans le cadre de leur formation initiale, d'une formation au monde du travail, aux professions et aux métiers. Cette formation spécifique me paraît particulièrement bienvenue. Elle doit aussi être l'occasion de former les enseignants et les cadres de l'éducation nationale aux enjeux de la digitalisation du monde en général, et de notre économie en particulier. Tel est le sens de l'ajout que je propose

de loi prévoit que les enseignants et les personnels d'inspection pourront être formés au monde économique et professionnel, ainsi qu'au fonctionnement des entreprises. Cette formulation assez large permettra de sensibiliser les enseignants aux différents enjeux auxquels sont confrontées les entreprises, dont ceux liés à la digitalisation.

il faut en effet qu'il y ait cette sensibilisation. Embarras, parce que je m'interroge sur l'intérêt de préciser cela au niveau législatif. On peut aussi penser à d'autres sujets non moins importants, comme la transition écologique, qui doivent également faire l'objet d'une sensibilisation.

Il ne s'agit pas de dire qu'ils ou elles n'ont pas leur place dans le dispositif d'accompagnement des jeunes, ce qui n'aurait aucun sens. Tout d'abord, ils participent au resserrement des options professionnelles les choix d'orientation lors de la scolarité. Orienter tel ou tel élève vers des options au lycée participe pleinement à la détermination d'un projet à long terme. Ensuite, les enseignants sont particulièrement bien placés pour donner des conseils d'orientation, étant au quotidien auprès des élèves. Toutefois, il ne me semble pas pertinent de surestimer ce rôle, car cela risquerait de dessaisir les conseillers d'orientation. Il serait préférable de recentrer les missions des enseignants sur l'instruction, plutôt que de miser sur leurs connaissances du monde économique et professionnel,

En effet, les formations professionnelles initiales, en particulier l'apprentissage, sont trop souvent méconnues, voire dévalorisées, et ne font pas l'objet de la promotion qu'elles méritent aux différentes étapes de l'orientation des élèves.

Il nous semble donc important que les actions de sensibilisation et de formation tiennent compte des enjeux liés au développement des nouvelles technologies, ainsi que des secteurs jugés à fort potentiel d'emplois sur le plan local, afin d'aborder de manière dynamique le monde économique et professionnel, les professions et les métiers. Cet amendement vise donc à préciser que ces formations devront prendre en compte les filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d'emplois aux niveaux tant régional que national. Il tend en que les formations destinées aux inspecteurs d'académie, aux inspecteurs pédagogiques régionaux, aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux chefs d'établissement, qui visent à améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, traitent également ces aspects.

en supprimant les mots « à portée régionale ». Cet alinéa prévoit que sont transférées aux régions et collectivités assimilées les missions des délégations régionales de l'ONISEP en matière de diffusion de la documentation, ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants. La notion de publications « à portée régionale » semble induire une distinction avec les publications à portée nationale au sein des délégations régionales de l'ONISEP. Quel est l'avis de L'alinéa 6 prévoit que la région élaborera avec le concours de l'ONISEP la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions. L'ONISEP demeurera compétent pour la documentation nationale. Par conséquent, il est utile de maintenir cette précision à l'alinéa 30, afin que soient transférées aux régions les missions à portée régionale. Cela permettra d'opérer un transfert de personnel cohérent de personnel cohérent avec cette nouvelle répartition des missions, dans le cadre des conventions de transfert qui seront conclues entre l'État et les régions. L'objectif, c'est que l'État et les régions se parlent.

Il s'agit de mieux préparer le transfert aux régions des missions exercées par les délégations régionales de l'ONISEP. De manière à le rendre cohérent avec la rentrée scolaire, cet amendement reporter le transfert en cause au 1 septembre 2019.

commission ? L'article 10 prévoit, d'une part, que la région élaborera, avec le concours de l'ONISEP, la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et les professions et, d'autre part, que ces missions à portée régionale, aujourd'hui exercées par les DRONISEP, seront transférées aux régions, ainsi que le personnel correspondant. Si une région ne demande pas ce transfert, deux éditeurs de documentation à portée régionale coexisteront : la région, au titre de sa nouvelle mission, et la DRONISEP non transférée. L'amendement n° 243 est donc de nature à complexifier le système.

Ce report donnera plus de temps aux régions pour s'approprier leurs nouvelles missions sur l'orientation et se concerter avec l'État pour assurer un transfert dans les meilleures conditions. Je suis donc favorable aux amendements

est la disposition essentielle du projet de loi qui doit permettre aux régions d'exercer pleinement leurs nouvelles compétences d'information des élèves et des étudiants sur les métiers et les formations. L'article 25 du texte précise que toutes les dispositions du titre I, ce qui inclut celles prévues à l'article 10,

à réguler les choses, car il y a déséquilibre. Soit il y a transfert de compétences, et on fait confiance aux régions, y compris pour avoir une vision nationale de l'orientation,

relève du même esprit. L'expérience des précédents transferts de compétences a montré que le délai de trois mois était souvent trop court. L'allongement du délai apparaît d'autant plus judicieux qu'en l'espèce quatre signataires sont prévus,

L'allongement du délai prévu pour signer la convention type de mise à disposition des services ou parties de services de l'État retardera la publication du décret de transfert définitif. Or le transfert aux régions des missions exercées actuellement par les délégations régionales de l'ONISEP est une disposition essentielle du projet de loi, parce qu'il doit permettre aux régions d'exercer pleinement leurs nouvelles compétences d'information des élèves et des étudiants sur les métiers et les formations.

chargé de coordonner les interventions des organismes participant au service public régional de l'orientation, à savoir les missions locales, le réseau CARIF-OREF, le réseau information jeunesse ... La loi 5 mars 2014, complétée par la loi du 27 janvier 2017, a confié aux régions la responsabilité de coordonner les actions de ces organismes, mais elles peinent à assurer ce rôle. Ces organismes continuent de recevoir des directives de leur ministère de tutelle, et les régions ne disposent pas des moyens que l'État leur affecte. L'amendement tend à prévoir que chaque comité disposera d'un conseil d'administration composé de représentants de la région, de l'État, des autres acteurs de l'orientation, des entreprises, ainsi que des parents d'élèves et des étudiants, la présidence du conseil d'administration étant assurée par le président du conseil régional ou son représentant. la commission ? L'adoption de cet amendement ouvrirait la possibilité aux régions de créer un comité régional de l'orientation avec l'État, afin de coordonner les différents acteurs du service public régional de l'orientation. Ce dispositif pourra être un outil utile de pilotage de l'orientation sur le territoire régional, que les régions pourront ou non mettre en place selon leurs besoins. L'avis est donc favorable. Quel est À mes yeux, la disposition proposée n'est pas nécessaire, le cadre juridique existant permettant déjà aux représentants de l'État et des régions de créer ce type d'agence pour renforcer la complémentarité entre Cela permet ainsi d'exercer plus efficacement la responsabilité dévolue aux uns et aux autres dans la coordination de l'action des organismes participant au service public régional de l'orientation. Il convient de préciser que la création d'une telle agence doit reposer sur un accord entre l'État et la région prévoyant, notamment, leurs contributions financières respectives. Mon avis est donc défavorable.

Ce faisant, le Gouvernement supprime aux régions des ressources qui finançaient, non seulement l'apprentissage, mais aussi, en partie, la formation professionnelle. Nous demandons ce rapport

Le scrutin est ouvert.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

Or, ce que chacun sait moins, c'est que les élèves de moins de quatorze ans n'ont le droit de faire leur stage que dans les administrations, les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales.

Puisque ce stage d'observation vise à faire découvrir aux élèves le monde professionnel et économique, à explorer les métiers et les formations et à développer leurs connaissances, il me paraît pertinent d'ouvrir le champ des possibilités et d'élargir la tenue de ces stages d'observation à toute entreprise régie par le droit privé. Bien entendu, comme le rappelle une note du ministère de l'éducation nationale, ce stage d'observation ne doit

La rédaction du code du travail est ambiguë et ne permet pas aux élèves de moins de quatorze ans, pourtant en quatrième, de faire ces stages en entreprise pendant les vacances scolaires. Nous soutenons donc cette clarification rédactionnelle visant à lever une interdiction qui n'est pas justifiée. La commission

Une telle possibilité est déjà ouverte aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, avec le soutien des chambres consulaires. Eu égard au succès rencontré par ces stages, qui permettent à de nombreux jeunes de découvrir des métiers, notamment ceux relevant du secteur de l'artisanat, et conformément au souhait exprimé par les organismes consulaires, le présent amendement vise à étendre ce dispositif aux étudiants des enseignements supérieurs. Quel Nous avons déjà débattu d'amendements similaires. Les étudiants ont déjà la possibilité d'effectuer des stages en milieu professionnel en dehors des heures de cours, sur la base d'une convention de stage entre leur université et la structure d'accueil.

Une année de césure permettrait aux étudiants d'obtenir, en plus de la licence, un CAP. Favoriser une plus grande perméabilité entre les différents univers professionnels permettra aux étudiants d'accéder à un plus grand nombre de débouchés sur le marché de l'emploi ainsi qu'à une double expertise. Les bénéficiaires de ces conventions n'auront plus à choisir entre un parcours universitaire et l'apprentissage d'un métier manuel. Cela permettra en outre de satisfaire leurs parents qui, souvent, s'opposent à leur orientation vers les CAP.

Les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent déjà demander à suspendre leurs études pour bénéficier d'une formation disjointe ou complémentaire de leurs études d'origine. La circulaire du 22 juillet 2015 du ministère de l'enseignement supérieur relative à la mise en oeuvre d'une période de césure

il n'apparaît pas opportun de limiter ce dispositif aux étudiants en licence et à la préparation d'un CAP, alors que tous les étudiants de la tranche d'âge peuvent prétendre à cette passerelle.

M. Max Brisson. Le campus des métiers et des qualifications a notamment des missions d'articulation entre la voie scolaire et la voie professionnelle. Les chambres consulaires ont un rôle renforcé en matière d'apprentissage. Il apparaît donc cohérent que ces entités participent aux campus des métiers et des qualifications.

et l'apprentissage, que le Gouvernement souhaite faciliter à travers le présent projet de loi. Il est indispensable que les centres de formation d'apprentis soient présents pour la réalisation de cet objectif. L'article 7 du présent projet de loi consacre les missions des chambres consulaires en matière d'apprentissage. Ces organismes sont donc des acteurs essentiels des politiques en faveur de l'apprentissage dans les territoires. Il convient de les intégrer au sein des campus des métiers. C'est donc un amendement de bon sens

satisfaits. L'article 10 prévoit que les campus des métiers regrouperont, notamment, des organismes de formation. Or les CFA deviendront des organismes de formation de droit commun en vertu de l'article 11 de ce

soit de lieux déjà existants, qui seront renforcés, soit de lieux nouveaux, en fonction des projets des régions, que l'État soutiendra au maximum. C'est d'ailleurs le sens des dialogues qui ont déjà commencé entre les régions et l'État, ce qui devrait nous rendre optimistes quant à la possibilité de cette cohérence entre l'État et les régions.

On peut espérer que les responsables de ces organismes sont au courant de la situation et qu'ils ont eu

issue du rapport d'Élisabeth Lamure sur l'apprentissage comme voie de réussite. Cette formation serait organisée par les centres de formation d'apprentis et permettrait une complète information des lycéens. Quel est l'avis de la L'article L. 313-1 du code de l'éducation pose le principe d'un droit au conseil en orientation et à l'information dans l'ensemble de l'enseignement scolaire. Il apparaît donc peu opportun de faire figurer parmi ces dispositions générales une mesure spécifique sur l'apprentissage et les missions des CFA, qui créerait en outre une contrainte non négligeable pour les CFA. Par ailleurs, les dispositions de l'article 10, que nous venons d'examiner, permettront de renforcer ce droit à l'information et à l'orientation et de faire découvrir aux élèves et étudiants les formations en apprentissage, notamment en association avec des CFA.

Ils peuvent le faire en partenariat avec les nombreux acteurs économiques locaux, que vous connaissez bien, madame la ministre, qu'il s'agisse des chambres de commerce, des missions économiques, des entreprises et filiales françaises ou des conseillers du commerce extérieur, qui sont susceptibles d'offrir des stages en entreprise.

J'aurais pu, d'ailleurs, y adjoindre un bon nombre d'autres acteurs économiques locaux. Nous avons tout à gagner à développer ce genre de filières, qui n'existent malheureusement pas. Nous avons en effet des classes préparatoires en fin de cycle, ne sont pas ouvertes à ceux qui ont d'autres compétences que celles qui leur permettent de suivre des études classiques. Par ailleurs, bon nombre de ces filières techniques

à Mme Laurence Cohen. Selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, à leur arrivée en CFA, certains jeunes maîtrisent mal des compétences essentielles à la vie sociale et professionnelle. La plupart d'entre eux ont fréquenté l'école durant durant une douzaine d'années et en gardent des acquis non négligeables, mais ils sont marqués par une relation difficile à l'univers de l'écrit, à celui des nombres et aux apprentissages scolaires. La réalité de l'illettrisme diffère selon les régions et selon les publics. En France, on estime que 7 % des personnes sont « illettrées » et 10 % des demandeurs d'emploi. Ce phénomène est loin d'être anodin tant par la suite les difficultés sont grandes pour trouver un emploi, une formation, remplir les démarches administratives du quotidien, etc. Loin de stigmatiser les personnes en situation d'illettrisme, l'évaluation des politiques régionales de lutte contre ce fléau proposée par la députée Béatrice Piron pourrait être un outil intéressant pour analyser les défaillances de notre système scolaire

c'est un outil important et essentiel qui permet le contrôle et l'évaluation des politiques publiques. En l'occurrence, seul l'État est en mesure de déployer la puissance nécessaire pour réaliser un état des lieux précis

réelles difficultés. Enfin, cela a été soulevé à plusieurs reprises, il est ici question du maillage du territoire et de l'accès à des services de proximité. Or les garanties qui sont données sur l'existence

est à Mme Catherine Morin-Desailly. Toutes les études et comparaisons internationales qui pointent du doigt les piètres performances des élèves français soulignent également l'insuffisance de la formation continue des enseignants, celle-ci revêt une grande importance dans des pays comme Singapour ou la Finlande, régulièrement en tête de classement. Or le code de l'éducation ne prévoit actuellement d'obligation de formation que pour les enseignants du premier degré.

à plusieurs reprises ces dernières années. Il me semble donc particulièrement utile de saisir l'occasion qui nous est donnée de marquer, par un signal fort, notre volonté en ce domaine. Bien entendu, d'autres réflexions seront engagées et des rapports

? Nous sommes d'accord sur le principe, mais la mise en oeuvre de ce dispositif risque d'être très compliquée et de représenter une charge considérable d'organisation pour le monde de l'éducation nationale, en particulier pour les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, compte tenu du nombre d'enseignants dont il faudrait assurer la formation continue. La commission souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement.

sont ceux vers lesquels les élèves se tournent immédiatement pour essayer d'obtenir des informations en matière d'orientation et pour mieux comprendre le système éducatif de l'enseignement supérieur. Or ils ne sont pas forcément formés à cela.

Mais l'histoire de notre commission est longue : cela fait plusieurs années que l'on travaille sur ce sujet et, à chaque fois, la question de la formation continue des enseignants

d'une part, en introduisant un financement au nombre de contrats et, d'autre part, en mettant en concurrence les formations. Cet article impose aux lycées professionnels et aux centres de formation de rendre publiques un certain nombre d'informations concernant leur fonctionnement le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels, le taux de poursuite d'études, le taux d'interruption en cours de formation, le taux d'insertion professionnelle à la fin de la formation et la valeur ajoutée de l'établissement. Transmettre de telles informations aux élèves et à leur famille sans les expliquer risque de les amener à juger les formations de manière biaisée. En effet, cet article prévoit de communiquer des données complètement déconnectées de la qualité d'une formation, telles que la valeur ajoutée d'une formation. formation. Si l'on veut être informé de la qualité d'une formation, il existe déjà des organismes chargés de cette mission, notamment les CIO, d'où l'importance de ne pas les fermer. Une autre mesure contribue à la mise en concurrence entre les filières d'apprentissage et les lycées professionnels : la possibilité d'ouvrir des filières d'apprentissage au sein des lycées professionnels. telle mesure a été déplorée par des directeurs d'établissement, qui craignent qu'elle soit source de violences. En effet, les étudiants des lycées professionnels sont en stage alors que les apprentis sont salariés. Deux élèves qui suivent pourtant la même formation peuvent donc recevoir des salaires très différents selon qu'ils sont en lycée professionnel ou en apprentissage. Ces mesures de mise en concurrence entre les centres de formation d'apprentis et les lycées professionnels tendent encore une fois à favoriser l'apprentissage, ouvert dès l'âge de quinze ans révolus. Or de si jeunes élèves devraient continuer à bénéficier du système d'éducation, et donc des lycées professionnels. La

que le contexte économique agricole actuel n'encourage déjà pas à la signature de contrats d'apprentissage dans un secteur soumis à de vraies spécificités- la saisonnalité des travaux, la soumission aux aléas climatiques, le caractère dangereux de certaines tâches, le travail avec des êtres vivants, le caractère coûteux du matériel. Rappelons-le, l'enseignement agricole est marqué par une territorialisation forte des cultures et des savoir-faire, la branche des métiers de l'agriculture n'est pas vraiment structurée et le deuxième pilier de la PAC est géré par les régions. Le projet de loi risque d'engendrer une désorganisation de l'enseignement agricole, d'autant plus à craindre en période de démographie décroissante. Une régulation par les branches semble illusoire, dans la mesure où celles-ci sont peu implantées dans les territoires.

Cet amendement vise à revenir sur l'une des dispositions qui introduisent une logique de marché dans le système d'apprentissage, notamment par l'instauration d'un financement des CFA lié au nombre de contrats conclus- ma collègue vient de le souligner. Actuellement, vous le savez, les CFA reçoivent une enveloppe globale, qui est complétée par d'éventuels financements, souvent importants, des régions. Cela permet de les développer de manière homogène, dans un souci d'équilibre et d'aménagement du territoire. Or la mise en place du financement par contrat revient, selon l'Association des régions de France, à la fermeture d'environ 700 CFA dans le pays,

centres, parce qu'ils sont dans des zones plus faiblement peuplées et dispensent des formations plus rares, des formations émergentes qui ne représentent pas de gros effectifs.

de supprimer cet article. Les CFA doivent pouvoir continuer d'exister dans la plupart de nos territoires ; c'est ce qui permettra à un maximum de nos jeunes d'accéder à des formations diverses et variées. Quel

pourront être librement créés, mais ils seront soumis au même régime de création et de déclaration d'activité que les organismes de formation. Ils resteront soumis à un contrôle pédagogique, ainsi qu'à un contrôle administratif et financier. En outre, des règles spécifiques sont prévues pour les CFA, compte tenu de leurs missions d'enseignement et d'accompagnement des apprentis, telles que des versements supplémentaires par rapport au coût des contrats.

France compétences n'aura pas la mission de publication des informations sur les formations des CFA et des lycées professionnels c'est le rôle des services de l'État- la DEPP, pour l'éducation nationale, et la DARES, pour le ministère du travail -, qui publient déjà des enquêtes sur le suivi des publics en alternance.

de contraintes de publication difficiles à assumer pour de petites structures. En outre, un effectif faible ne permettra pas de dégager des données objectives sur la qualité du CFA ou du lycée professionnel-

L'Assemblée nationale a ajouté, parmi les informations que devront communiquer chaque année les centres de formation d'apprentis et les lycées professionnels, la « valeur ajoutée » de leur établissement. Le présent amendement vise à supprimer ce critère, totalement imprécis et non évaluable.

Les établissements pourront avoir du mal à appliquer cette obligation. Par conséquent, il sera compliqué d'effectuer une évaluation comparée des établissements sur cette notion imprécise. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement. Quel est

La durée minimale d'un apprentissage sera ramenée à six mois ; un minimum de 150 heures de période d'apprentissage semble donc satisfait. La modulation de la durée minimale pourra intervenir pour prendre en compte les acquis préalables de l'apprenti,

Magner. Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat, qui confie la présidence du conseil d'administration des lycées professionnels à l'une des personnalités extérieures qui le composent. Plus grave encore, il suffirait qu'il y ait, dans l'établissement, une section d'enseignement professionnel pour que cette règle s'impose. Je le sais, le conseil d'administration des lycées agricoles est présidé par des personnalités extérieures, mais il s'agit d'un type spécifique d'établissement et d'enseignement, qui relève d'ailleurs du ministère de l'agriculture et non de celui de l'éducation nationale. Un bon chef d'entreprise n'a pas forcément de grandes qualités de pédagogue ni de connaissance de l'ensemble des enseignements ; il n'aura pas forcément l'écoute ni la confiance de l'ensemble du corps professoral. En outre, que penser de la situation d'un lycée d'enseignement général qui comprendrait une section d'enseignement professionnel et qui serait alors présidé par un chef d'entreprise et non par son proviseur ?

Il est, selon nous, indispensable que les lycées professionnels se rapprochent du monde économique et professionnel. C'est pourquoi la commission a souhaité confier la présidence du conseil d'administration des lycées professionnels à une personnalité extérieure, qui pourra être issue du monde de l'entreprise.

ni un argument ni une référence. On le lui dira ! Chacun peut trouver des témoignages qui lui conviennent, comme chacun est capable de trouver des citations qui confirment la philosophie qu'il développe. Il y a tout de même dans ce que vous dites un danger et- veuillez m'excuser, je ne trouve pas d'autre mot -une forme d'hypocrisie. Nous laisser entendre qu'il pourrait y avoir à la tête d'un établissement un président qui ne servirait à rien et un proviseur qui, lui, aurait toute latitude pour conduire non seulement la pédagogie, mais encore l'organisation de son établissement- la pédagogie est sérieusement dépendante de l'organisation, du projet d'établissement -signifierait que l'on a un président complètement fantoche.

vote. Il n'y a pas que des lycées professionnels publics, il y a aussi, par exemple, des lycées professionnels privés sous contrat d'association. Il ne faut pas confondre le rôle du chef d'établissement et celui du président du conseil d'administration.

Cet amendement de clarification vise à éviter une incohérence avec les attributions du président du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement ce dernier ne disposant pas de pouvoir décisionnaire, il ne peut donner un accord. Sa seule attribution est de présider les séances du conseil d'administration ; les unités de formation par apprentissage seront donc créées sur l'initiative du seul chef d'établissement.

Il s'agit de sécuriser les parcours d'orientation des personnes en situation de handicap, qui rencontrent en effet de nombreuses difficultés pour s'inscrire dans un parcours d'apprentissage. Pour développer l'accès à l'apprentissage, en particulier des jeunes handicapés, il convient que les CFA s'adaptent à leurs besoins. Nous devons avoir une politique volontariste pour cela. Tel est le sens de cet amendement. De nombreux aménagements sont déjà prévus pour les apprentis en situation de handicap, qu'il s'agisse de l'exécution du contrat d'apprentissage, de sa durée ou encore des obligations de l'employeur. En outre, l'article 11 renforce l'accompagnement des personnes handicapées parmi les missions des CFA. Chaque CFA devra désigner un référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap. Il ne paraît pas nécessaire

assistent » les postulants dans leur recherche d'apprentissage. Or ces centres sont en relation constante avec les entreprises et les professionnels ; ils sont donc les mieux placés pour évaluer les besoins, les attentes et les capacités des deux parties

sur celui des offres de stage en université- recensement et accompagnement. Les CFA pourraient en effet, je le répète, participer plus activement à la recherche des contrats d'apprentissage pour renseigner les postulants et les orienter en fonction de leurs aspirations et de leur CV.

Les CFA auront pour mission d'assister les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur. En pratique, leur connaissance des entreprises locales leur permet déjà d'accompagner efficacement les candidats dans la conclusion de leur contrat d'apprentissage. Nous

? Les CFA peuvent déjà accueillir des personnes en période de mise en situation en milieu professionnel, mais il est utile de le préciser clairement dans leur mission,

L'apprentissage, dans l'enseignement agricole, est en grande majorité dispensé dans des centres publics, les CFAA, avec 205 sites publics et 75 % d'apprentis formés. Les CFAA et leurs antennes constituent un maillage fort du territoire, du fait de leur implantation en zones rurales, où pèse la désertification des services publics, d'autant qu'ils comportent des exploitations ou des ateliers pédagogiques au service des élèves, apprentis, stagiaires et étudiants, en lien avec le tissu économique local. Ils dispensent des formations avec des effectifs parfois inférieurs à 10 apprentis, qui sont parfois des jeunes peu mobiles et éloignés des parcours sociaux et professionnels conventionnels. C'est pourquoi il convient de reconnaître dans le chapitre du code du travail relatif aux missions et obligations des CFA la spécificité des centres Madame la ministre, vous n'êtes pas sans connaître les craintes et les risques que ce projet de loi, associé à la réforme du lycée, fait naître au sujet de la filière d'enseignement agricole public, puisque vous avez reçu très récemment- c'était le 6 juillet dernier -les représentants d'une intersyndicale. La presse s'est fait l'écho

son rôle dans la démocratisation de l'accès aux diplômes, pour que nos jeunes puissent continuer à vivre dans nos territoires ruraux. Nombre de structures à la taille modeste et aux effectifs réduits, caractéristiques qui participent, d'ailleurs, à la réussite de cet enseignement spécifique, ne sont pérennisées que grâce au soutien régional, que le financement par les seules branches professionnelles viendrait remettre en cause. Cet amendement est donc un amendement d'appel en faveur du maintien et de la protection des formations de l'enseignement agricole public et, en premier lieu,

Nous comprenons le sens de cet amendement d'appel. Tous les membres de la commission des affaires sociales sont attachés à la formation en apprentissage dans le domaine agricole et au maintien des centres de formation en zone rurale. Toutefois,

au titre de l'aménagement du territoire. La commission a également complété les critères à retenir pour le coût au contrat, qui devra tenir compte des apprentis résidant en zone rurale. C'est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

apprenti. D'ailleurs, les secteurs qui sont très dynamiques en matière d'apprentissage- je pense notamment à l'agriculture et à l'artisanat -bénéficieront beaucoup plus qu'aujourd'hui de la péréquation,

afin d'offrir aux personnes en situation de handicap les mêmes outils d'apprentissage et de meilleures capacités d'insertion professionnelle. C'est un dossier très important, dont nous aurons l'occasion de reparler au titre

cet amendement incitera les développeurs de logiciels et de progiciels à créer des outils numériques, qui, dès leur conception, sont natifs, accessibles. Il s'agit là d'une exigence démocratique, qu'il nous faut inscrire dans la loi pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle, l'autonomie et le maintien dans l'emploi des apprentis en situation de handicap. Cette exigence est d'autant plus légitime que les métiers du numérique représentent un secteur très adapté aux futurs travailleurs handicapés. En favorisant l'accessibilité universelle et originelle des outils numériques, on améliore, dans le même temps, la formation initiale et l'insertion professionnelle. Quel est l'avis de la ? Le code du travail prévoit déjà des aménagements pour l'accessibilité aux personnes handicapées des outils pédagogiques utilisés en CFA. Par ailleurs, cet amendement ne vise que les cas dans lesquels des enseignements normalement dispensés par des CFA sont assurés par des établissements d'enseignement. La commission est donc défavorable

par les prestataires de formation soumis à l'obligation de transmission d'un bilan pédagogique et financier. Cet accès permettrait d'affiner l'expertise de France compétences s'agissant des coûts de formation, en complétant l'accès aux informations transmises aux organismes financeurs par les prestataires de formation, prévu à l'article L. 6353-10 du code du travail, et lui permettrait de bénéficier du même droit d'information que celui des opérateurs de compétences pour ce qui concerne les centres de formation des apprentis, lequel figure à l'article L. 6351-7 du même code. La transmission de ces documents par les organismes de formation à l'autorité administrative est destinée à assurer le contrôle pédagogique administratif et financier de ces organismes. France compétences n'exercera pas cette mission. S'agissant de la mission de péréquation pour les formations en alternance attribuée à France compétences, un décret en Conseil d'État en précisera les modalités d'application, comme le prévoit l'article 16.

Mme Monique Lubin. Madame la ministre, nous pensons que votre réforme fait peser de nombreux risques sur les CFA, tout particulièrement durant la phase de transition vers le nouveau système de financement. Les CFA les plus fragiles doivent être sécurisés d'un point de vue financier. C'est la raison pour laquelle nous proposons que le dispositif transitoire d'affectation des éventuels excédents de taxe d'apprentissage au titre de l'exercice 2019 prenne en compte les éventuels déficits des CFA après certification par un commissaire aux comptes, du fait, par exemple, d'une insuffisance de taxe d'apprentissage au regard du nombre d'apprentis formés. Avant de basculer dans le financement par contrat d'apprentissage, les CFA doivent disposer d'un minimum de trésorerie pour fonctionner pendant la période transitoire. Au titre de sa mission de péréquation, il peut être utile que les excédents de taxe d'apprentissage récupérés par France compétences servent à couvrir les éventuels déficits des CFA sur l'année 2019, afin qu'ils basculent dans le nouveau système de financement « au contrat

cet amendement. En effet, ce n'est pas la trésorerie des CFA qui va être reversée à France compétences : ce sont les reports de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire de l'apprentissage au titre du dernier exercice. Les CFA vont donc bien garder leur trésorerie ordinaire pour pouvoir

La possibilité de créer librement des CFA, à titre dérogatoire, dès la publication de la loi, alors même que le nouveau régime ne sera pas encore mis en place, doit être accompagnée de garanties. À ce stade, nous disposons de peu d'informations sur cette dérogation, qui a été introduite à l'Assemblée nationale. Il peut être risqué de faire coexister deux régimes juridiques pour les CFA pendant la période transitoire.

non pas une dérogation accordée à de nouveaux organismes de formation, mais simplement l'application de la loi entrée en vigueur. La création d'un nouveau CFA nécessitera une déclaration, puis une certification dans les dix-huit mois qui suivent.

Le scrutin est ouvert.

213. Cet amendement fait partie d'un tout où figure la question des dispositifs de préapprentissage, mais aussi celle de l'orientation.

à mi-chemin entre le lycée professionnel et l'usine », comme l'écrivait le journal en avril dernier. On ne peut le nier, du côté des familles, c'est surtout le soulagement qui prime, car les 800 élèves formés chaque année ont souvent pour point commun une situation scolaire en péril et un risque de Ce dispositif constitue en quelque sorte une autre forme d'apprentissage. Quel en est le concept ? Les élèves restent dans l'établissement en permanence et consacrent les deux tiers de leur temps à remplir des commandes d'entreprises locales et à produire pour ces mêmes entreprises. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant que ce soit bien plus souvent des foyers économiques locaux qui poussent à l'ouverture d'écoles de production. Ce système s'expose toutefois à des dérives en

si le Parlement va au bout de la reconnaissance législative des écoles de production, quelles seront les conséquences pour l'apprentissage et pour le lycée professionnel ? Une entreprise n'aurait plus aucun intérêt à accueillir ces jeunes, puisqu'elle pourrait tout simplement passer commande auprès des écoles de production.

introduit cet article selon lequel les universités devraient créer des filiales de droit privé pour valoriser leurs filières professionnelles.

les gains financiers dégagés par la formation continue dans l'université ne pourraient plus être reversés au pot commun des UFR. Ils resteraient dans le giron de la formation continue, alors que les locaux, les personnels administratifs,

afin de dégager des revenus supplémentaires. Ces établissements accomplissent une mission de service public. Leur offre de formation ne doit pas être dictée par la recherche de profits. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

les convaincre de franchir le pas de l'apprentissage. Cette aide deviendra alors un dispositif supplémentaire de réduction du coût du travail. Je ne cherche pas opposer les TPE aux PME, mais il y a fort à parier que ce sont les structures les plus efficaces en termes de recherche de subventions qui en profiteront majoritairement,

en rassemblant les dispositifs existants dans un seul creuset, vous gommez les aides spécifiques aux travailleurs handicapés, déjà peu nombreux en apprentissage. En renvoyant à un décret ultérieur du Conseil d'État la mise en place des aménagements pour ces travailleurs, vous finissez de les exclure définitivement du dispositif. Il nous semble indispensable de maintenir l'accompagnement de l'État pour les entreprises. Toutefois, ce soutien doit chercher à corriger les effets du marché,

L'ensemble des acteurs auditionnés par vos rapporteurs se félicite de la simplification que constituera la fusion des aides aux employeurs d'apprentis. Les moyens budgétaires alloués aux précédentes aides seront reconduits au profit de cette nouvelle aide aux entreprises, soit environ 700 millions d'euros. En outre, les exonérations de cotisations sociales seront maintenues, ce qui représente 1,2 milliard d'euros d'allégement de charges pour les entreprises recrutant des apprentis.

pour les contrats d'apprentissage préparant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle au-delà du baccalauréat. Circonscrire l'aide aux diplômes et titres de niveau équivalent au baccalauréat aurait pour effet de limiter le développement de la qualification des jeunes, qui auraient plus de difficultés pour trouver une entreprise d'accueil. De plus, la mesure visant à limiter l'aide au niveau du baccalauréat apparaît incohérente avec celle visant à reculer l'âge maximum d'entrée en apprentissage à vingt-neuf ans révolus, les candidats à l'apprentissage les plus âgés ayant de fortes chances de viser les diplômes de niveau plus élevé.

Ces amendements visent à limiter l'aide unique aux entreprises de moins de 50 salariés, alors qu'elle est prévue jusqu'à 250 salariés par le texte. Il faut certes soutenir les TPE, mais aussi les PME qui doivent développer l'apprentissage. Les petites entreprises seront déjà soutenues avec l'aide prévue. En outre, il est préférable de concentrer l'aide sur les apprentis de niveaux IV et V, dont le recrutement est beaucoup plus difficile pour les employeurs.

n° 166 rectifié,

Mme Sabine Van Heghe. Cet amendement vise à sécuriser le dispositif d'aide aux employeurs d'apprentis en situation de handicap et à permettre au CNCPH d'avoir un droit de regard sur les aménagements prévus par le décret.

: La parole est à M. Daniel Chasseing. Le présent amendement vise, en complément des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre du plan Étudiants, à élargir à l'ensemble des niveaux de qualification les conditions d'accès au crédit d'impôt apprentissage. Celui-ci bénéficie aux entreprises qui embauchent un apprenti en première année d'apprentissage. En effet, afin d'encourager la poursuite des études entre le secondaire et le supérieur, comme le développement de l'offre de formation, tout en préservant la spécificité de l'apprentissage,

Nous défendons le choix de fusionner les aides afin de simplifier les démarches des entreprises. Maintenir le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage et élargir ses bénéficiaires reviendrait à diluer les moyens alloués au soutien des entreprises qui emploient des apprentis.

Toutefois, circonscrire la nouvelle aide unique à celles qui concluent des contrats d'apprentissage au niveau bac ou infra-bac va à l'encontre du discours de valorisation porté par le Gouvernement. Il importe valorisation porté par le Gouvernement. Il importe de casser la culture de l'échec qui est associée à l'orientation en apprentissage avant le baccalauréat. Il faut également continuer à développer l'apprentissage dans les niveaux supérieurs, qui pourra à la fois nourrir une culture de l'entrepreneuriat et entretenir la réputation d'excellence ayant vocation à caractériser toutes les formations en alternance. Très bien ! Quel est l'avis de la

Max Brisson. Toutes les mesures facilitant le recours à l'apprentissage sont les éléments intéressants de ce projet de loi. Elles permettent de corriger un certain nombre d'erreurs qui ont pu être commises, en particulier depuis 2012. 2012. Nous proposons d'aller plus loin et d'exonérer de toute cotisation et contribution sociales l'entreprise, quelle que soit sa taille, qui embauche en contrat d'apprentissage son premier apprenti, et ce pendant la durée du contrat. Quel est l'avis de la ? Je fais remarquer au préalable que les entreprises de moins de 250 salariés peuvent déjà recevoir une prime d'au moins 1 000 euros au titre de l'aide au recrutement d'un premier apprenti ou d'un apprenti supplémentaire, en application de l'article L. 6243-1-1 du code du travail. L'objet de l'article 12 est de fusionner en une aide unique quatre dispositifs actuels, à savoir deux primes régionales, une prime pour l'emploi d'apprentis handicapés et un crédit d'impôt. En outre, il existe déjà des règles d'exonérations de charges sociales pour les entreprises qui accueillent des apprentis. Les entreprises de moins de onze salariés sont ainsi exonérées de toutes les cotisations pour les salaires versés aux apprentis, professionnelles. Je pense qu'il est préférable de ne pas créer un nouveau dispositif de soutien au moment même où l'on veut rationaliser les aides à l'apprentissage.

Nous abordons l'examen d'un nouveau dispositif introduit par amendement à l'Assemblée nationale : la reconversion ou la promotion par alternance. Ce dispositif est destiné aux salariés en CDI ou en contrat unique d'insertion souhaitant changer de métier ou de profession ou bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle. Ils utiliseront pour cela les actions de formation dont l'objet est identique aux actions d'apprentissage ou de formation dispensées dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Une question se pose concernant les bénéficiaires. Le dispositif prévoit en l'état que seuls les salariés ayant un certain niveau de qualification seront concernés, ce qui vise les salariés les moins qualifiés. Toutefois, nous ignorons quel sera le plafond fixé par décret et ne disposons pas d'étude d'impact.

La mise en place de ce système de promotion ou de reconversion par alternance fait suite à un constat que nous faisons tous : nous allons au-devant de mutations très profondes du marché du travail.

des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes selon la taille de l'entreprise. Ce dispositif prévoit que les entreprises s'engagent à conserver les mêmes salariés,

que nous venons d'examiner. Il convient d'ouvrir à tous les salariés en CDI, quel que soit leur niveau, le bénéfice du nouveau dispositif de reconversion ou de promotion par alternance. Les parcours de reconversion ou de promotion sont susceptibles

à Mme Laurence Cohen. L'article 13 de ce projet de loi contribue à faire reposer sur le salarié la responsabilité de se former pour être être plus employable. Pour commencer, il tend à supprimer la possibilité laissée aux salariés et aux employeurs de convenir d'une prise en charge de la formation par l'entreprise, lorsque la durée de la formation souhaitée dépasse le nombre d'heures disponibles sur le CPF du salarié. telle disposition risque de limiter la possibilité pour les salariés de recourir à des formations longues. Seuls les salariés pouvant financer la part excédentaire de la formation Cette mesure paraît paradoxale compte tenu des ambitions du Gouvernement, qui sont de « développer les droits individuels des salariés » et de les rendre « concrets et réels

D'abord, cette obligation incombe à l'employeur et non à Pôle emploi. Ensuite, l'objectif de la formation continue doit être de permettre aux individus d'acquérir des diplômes et des qualifications valables sur l'ensemble du territoire, voire au niveau de l'Union européenne. En effet, la qualification permet d'attacher aux personnes des capacités à tenir des postes de travail de manière générale, tandis que les compétences ne sont que des apports supplémentaires mobilisables dans des situations particulières. Comme dans de nombreuses autres dispositions de ce projet de loi, le rôle de la formation professionnelle est détourné.

le dire au sujet de l'amendement précédent, le droit en vigueur prévoit déjà, pour les demandeurs d'emploi, que le contenu de la formation est défini par l'employeur en concertation avec Pôle emploi et l'OPCA, qui deviendra OPCO. Par conséquent, l'entreprise intéressée est déjà impliquée, et les branches pourront, plus généralement, faire part de leurs besoins en compétences auprès de leur opérateur de compétences. Il n'est donc pas nécessaire de remplacer l'OPCO par la branche.

Dans les faits, cette suppression brutale au profit de la logique d'individualisation du CPF va déstabiliser de nombreuses entreprises et se fera au détriment de l'évolution professionnelle et du maintien dans l'emploi des salariés les moins qualifiés. Il est donc proposé de prolonger le dispositif jusqu'à la fin de l'année 2018, afin d'assurer le financement des périodes intégrées dans les plans de formation pour 2018 et d'aménager une période de transition qui laissera aux entreprises les moyens d'adapter leur politique de professionnalisation.

31 décembre 2018. Or l'article 25 du projet de loi prévoit déjà que le titre I, relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage, entrera en vigueur au 1 janvier 2019. Le tuilage existe donc

professionnalisation-inclusion » dans un périmètre plus large, ouvert aux demandeurs d'emploi de bas niveau de qualification et réservé à certains employeurs, en particulier du secteur non marchand ou d'intérêt collectif. Ce dispositif permettrait de renforcer la formation

L'amendement n° 103 rectifié est satisfait par un amendement déjà adopté par l'Assemblée nationale, qui a permis de faciliter le recours aux contrats de professionnalisation pour les structures d'insertion par l'activité économique-

En outre, le texte prévoit déjà une expérimentation afin que le contenu de la formation soit défini par l'entreprise et par l'opérateur de compétences. L'accès aux contrats de professionnalisation est également facilité pour les structures par l'insertion économique. Par conséquent, expérimenter une nouvelle catégorie de contrats de professionnalisation, uniquement centrée sur le secteur non marchand, risquerait de brouiller un paysage qui